La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Le courage et l'abnégation dont les victimes de violences au sein de l'école de Saint-Cyr ont fait preuve, en témoignant et en dénonçant les exactions subies de manière organisée, doivent être suivis par une politique volontariste d'élimination des risques. Dans le cadre de la cellule Thémis, le ministère des armées doit ainsi poursuivre un travail de sensibilisation, d'information et de formation pour permettre aux victimes de témoigner. Il doit également poursuivre et accroître son travail d'écoute et d'accompagnement spécifique des victimes. La cellule Thémis produit un rapport d'activité annuel, ainsi que différentes statistiques, qui sont diffusées auprès des armées et des services. Quatre types de statistiques doivent figurer au sein du bilan annuel : celles qui relèvent des dossiers ouverts, celles qui concernent les dossiers en cours de traitement, traités ou archivés, celles qui visent les cas de harcèlement, discrimination et violence sexiste ou sexuelle et, enfin, celles qui portent sur les victimes et auteurs présumés.

Le ministère est ainsi invité à poursuivre son travail d'observation et d'élaboration de statistiques, pour mieux connaître la réalité des cas de harcèlements, de discriminations et de violences sexuelles ou sexistes au sein du ministère des armées et prendre ainsi les mesures nécessaires à l'optimisation de la cellule Thémis et,, à l'éradication des violences sexistes et sexuelles au sein des armées.

Il s'agit de leur fournir un uniforme évolutif pour toute la période de la grossesse. En effet, aujourd'hui, on relève une inégalité dans la tenue vestimentaire entre les femmes et les hommes, qui pénalise de fait les femmes militaires, obligées de porter une tenue civile sans distinction de grade. Or, ces différences ne sont pas sans incidence dans un milieu aussi hiérarchisé que la profession militaire. Cela n'aide pas à améliorer la manière dont sont considérées les femmes dans l'institution. Depuis 1970, la modification du statut des militaires confère les mêmes droits et obligations aux femmes et aux hommes militaires. Depuis 1975, le port de la tenue militaire est possible pour les femmes et oblige leurs collègues à les appeler par leur grade, et non plus par « madame » ou « mademoiselle ».

Je tiens à souligner qu'il ne faut pas voir dans cette disposition une obligation : aujourd'hui, la tenue civile est autorisée et, si elle est jugée plus confortable, elle peut bien sûr continuer à être portée.

à vous remercier

à l'action du ministère en matière de lutte contre les discriminations selon les origines, l'objectif étant d'encourager la diversité à tous les postes et grades. Après les récents cas de harcèlement et d'agression sexuelle, notamment à l'école militaire

En effet, pour faire évoluer leurs compétences et maintenir une culture de l'innovation dans un secteur qui se caractérise par une évolution technologique très rapide, les ingénieurs ont besoin de mobilité durant leur carrière. Il est donc nécessaire qu'ils puissent effectuer des allers-retours entre le secteur privé et la DGA.

Néanmoins, dans le cadre d'emploi effectif ou doctrinal, les réserves ne sont pas utilisées comme des unités organiques collectives véritablement combattantes. Cette acquisition de compétences nouvelles pour les réservistes, mais non pour les unités dont ils dépendent, se fera à coûts raisonnés,

Toutefois, s'il ne faut pas sortir l'armée du giron républicain- telle n'est pas mon intention -, il me semble essentiel de rappeler que, depuis la généralisation de l'instruction scolaire, c'est en priorité l'école qui est garante de la formation citoyenne des jeunes. annexé marque un retour en arrière problématique, qui s'inscrit totalement dans la volonté de mettre en place un service national universel. on transfère ainsi le lien entre la République et les citoyens de l'école vers l'armée. Or l'école est encore le lieu de la connaissance, de la culture, de l'apprentissage, du partage et du développement de l'esprit critique. Tout cela façonne la citoyenneté,

Nous souhaitons tous un meilleur avenir pour nos jeunes. Donnons-nous-en les moyens humains et financiers ! Des jeunes restent à l'écart de ces structures : échec scolaire, précarité de nombreux étudiants, chômage, parents en difficulté, etc.- vous connaissez le tableau aussi bien que moi,

Avant même le bilan qui interviendra à la fin de 2018, il existe déjà un consensus sur la valeur ajoutée de l'existence de ce dispositif. Cet amendement tend à s'assurer de sa consolidation, même dans la perspective de la mise en place du service national universel, le SNU, puisque celui-ci n'entraînera pas la suppression du SMV. de ce que l'on en sait, ils n'ont pas les mêmes finalités. S'il est un premier contact avec l'armée, le SMV ouvre à tous un dispositif d'intégration et de formation aux métiers proposés par l'armée, ce qui ne sera manifestement pas la vocation du SNU.

Cette première expérience donne l'occasion d'accueillir un peu plus de 2 000 jeunes. Pratiquée par des partenaires diversifiés- entreprises, services publics, hôpitaux, associations, collectivités territoriales -et destinée à des jeunes en très grande difficulté, ceux que l'on appelle du nom étrange de « décrocheurs

du Gouvernement ? Madame la sénatrice, vous faites bien de mettre en lumière le service militaire volontaire, qui est un très beau dispositif, vous l'avez dit,

comme un acteur incontournable de la politique du ministère des armées à destination des jeunes. La commission est en fait un lieu unique de dialogue entre le ministère des armées et la société civile. Centre de réflexion sur les questions relatives aux jeunes et aux armées, elle est un organisme de proposition à l'intention du ministre des armées et une structure opérationnelle d'action au profit des jeunes- contrat armées-jeunesse, prix armées-jeunesse, journées sport armées-jeunesse et des événements autour de thèmes à caractère éducatif ou mémoriel. est aussi la seule commission de ce type qui subsiste, et nous sommes conscients que son rôle doit faire l'objet d'une redéfinition pour l'adapter aux réalités de la jeunesse du XXI siècle. Le sujet nous paraît donc essentiel, et c'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement. Quel est l'avis de la

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que l'alinéa proposé soit inséré après l'alinéa 274.

Delattre. Le rapport annexé rappelle que le lien entre la jeunesse et les armées constitue un enjeu essentiel de la cohésion nationale et énumère les vecteurs contribuant à son affermissement. Comme vous le savez, mes chers collègues, le service civique attire de plus en plus de candidats. Ce sont déjà près de 270 000 jeunes qui ont effectué une mission. Le RDSE, attaché au service civique qu'il a contribué à instaurer en 2010, souhaite que cet engagement soit mentionné également comme un outil de rapprochement entre les armées et la jeunesse. En effet, parmi les missions citoyennes proposées au titre du service civique, certaines concernent aujourd'hui la défense. L'année dernière, l'armée de l'air a ouvert ses portes à des jeunes en service civique sur des bases aériennes situées dans l'hexagone et outre-mer. Cette année, elle accueille encore une trentaine de candidats. Par ailleurs, certains jeunes ont exercé au sein de collectivités locales, pour la restauration de lieux de mémoire.

parole est à Mme Hélène Conway-Mouret. Dans le cadre de cette nouvelle loi de programmation militaire, les dépenses destinées à la dissuasion nucléaire vont pratiquement doubler entre 2019 et 2025. Elles passeront d'une moyenne annuelle de 3,2 milliards d'euros, entre 2014 et 2019, à 5 milliards d'euros entre 2019 et 2023, et approcheront les 6 milliards d'euros en 2025. C'est un choix politique assumé, qui s'inscrit dans la continuité de décisions qui ont été prises par les gouvernements successifs et qui ont été garantes de notre paix jusqu'à présent. Sur un sujet très important lié à notre sécurité et, surtout, à la défense du territoire, face à l'évolution d'un monde dans lequel les rapports de force changent rapidement, mais aussi lorsque l'on voit comment, aujourd'hui, des acteurs mondiaux majeurs bousculent la notion même de dissuasion, il nous paraît opportun d'organiser un débat au niveau national sur cette question, afin d'informer et de sensibiliser nos concitoyens. Il ne s'agirait en aucun lieu d'un sondage ni même d'un référendum. Ce serait une occasion pour les Français d'être correctement informés et de s'approprier le thème du nucléaire militaire au travers d'un débat porté, par exemple, par les parlementaires. Je sais combien le Gouvernement est sensible à l'idée de lancer des débats, comme le montre l'exemple de la consultation citoyenne qui vient d'être lancée sur l'Europe. Ce débat pourrait être porté par le Parlement et répondre ainsi aux besoins des populations locales directement concernées par le dispositif français de dissuasion nucléaire.

une demande qui a été formulée au cours de ce débat par la Haute Assemblée et à laquelle je m'étais engagée à répondre favorablement. Nous touchons, en effet, à l'une des pierres angulaires de la présente loi de programmation militaire. Dans ce rapport annexé, à l'alinéa 349,

à horizon de 2030. J'ai en effet eu l'occasion, notamment lors des auditions en commission, d'expliquer que nous étions partis d'un travail de projection à 2030, pour pouvoir nous figurer ce que devrait être un modèle d'armées complet.

mentionne également la situation du parc en 2019, c'est-à-dire au démarrage de la loi de programmation militaire. On voyait, dans la version initiale, le parc à la fin 2025. Or vous avez souhaité pouvoir disposer d'un point d'information à horizon de 2021, qui est la date à laquelle nous aurons notre rendez-vous, afin de pouvoir procéder à l'actualisation de la loi de programmation militaire en vue de sécuriser la réalisation de l'objectif de 2 % du PIB en 2025. Cet amendement me paraît donc répondre très directement à la demande que vous aviez formulée. Il permet, par exemple, de constater que, sur les SNA, les sous-marins nucléaires

2021. Je crois avoir répondu à une demande extrêmement forte de votre Haute Assemblée.

à une position qui n'était pas celle que nous avions initialement imaginé tenir. Nous avons en effet émis un avis favorable 30 d'entre eux. Nous avons également réprimé notre première intention, qui eût été de donner un avis défavorable, pour 32 d'entre eux, et nous nous sommes ralliés

Cela demandera un glossaire en complément de tous vos tableaux, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles pour le commun des mortels ... Naturellement, je voterai cet amendement. Je voudrais en profiter, si vous me le permettez et sans aucune flagornerie,

l'honnêteté de reconnaître que le Sénat avait été utile pour cette loi de programmation militaire, je ne doute pas que vous compterez sur la Haute Assemblée et que vous ne manquerez pas de l'écouter lorsqu'il s'agira de traduire cette loi, à l'occasion des différents votes annuels qui vont concrétiser la bonne volonté que nous avons tous manifestée. Je

Conway-Mouret. Madame la ministre, cet amendement a pour objet d'attirer votre attention sur la nécessité d'assurer le maintien d'une capacité de production industrielle de composants stratégiques sur notre territoire. Or cette production repose, pour une bonne part, sur un tissu de PME françaises. pays dispose, en effet, hormis ses dix grands groupes industriels, de multiples petites et moyennes entreprises- près de 4 000 -engagées dans la production industrielle du secteur de la défense. Nous en avons tous sur nos territoires. Nous devons les protéger et les promouvoir, car, si l'intention du Gouvernement est de développer « des politiques de long terme en matière de recherche, d'investissement, de protection du potentiel scientifique et technologique français », il est illusoire d'espérer y parvenir sans une base de production industrielle importante et performante sur notre territoire. C'est particulièrement important pour l'ensemble de la chaîne de production des composants de matériels de défense. Seule une politique industrielle performante sur notre territoire même, qui encourage la formation d'emplois qualifiés, développe des infrastructures et soutient la modernisation des outils de production, permettra de développer la recherche et le développement dont nous avons besoin pour assurer notre autonomie stratégique. Nous devons ainsi protéger ces PME. La protection de leur capital industriel et intellectuel par l'État est une nécessité, afin d'en éviter le pillage et de permettre leur développement économique, notamment dans la recherche de fonds, indispensable au financement de leurs efforts de recherche et de développement. Nous souhaitons, par cet amendement, que cette dimension et ce souci de protection de nos PME liées à l'industrie de défense puissent être pris en compte à l'alinéa 378 de l'article 2 de ce projet de loi. Quel Nous approuvons, bien évidemment, la volonté, soulignée par cet amendement, de maintenir les capacités technologiques, les capacités d'innovation, les capacités industrielles de nos entreprises sur le territoire national.

faut permettre à nos entreprises de s'affronter à nos concurrents internationaux ! Pour ce faire, peut-être faudrait-il revoir notre fiscalité et la façon dont on appréhende notre outil de compétitivité industrielle. Aujourd'hui, tout a basculé à cause

et fasse référence aux programmes engagés et à venir avec tous les acteurs et partenaires principaux de la France. Si l'on se réjouit de la volonté de travailler en coopération avec l'Allemagne, il faut souligner que, jusqu'à présent, notre partenaire privilégié a été le Royaume-Uni, notamment dans les OPEX. Le processus du Brexit ne doit pas empêcher de continuer à coopérer en matière de sécurité et de défense, car de nombreux programmes relèvent d'accords bilatéraux déjà en place. La revue stratégique promet d'ailleurs le maintien d'un lien bilatéral solide avec le Royaume-Uni, d'une coopération « structurante ». Elle insiste sur la nécessité « de maintenir une relation de défense privilégiée avec le seul pays européen toujours doté d'ambitions globales, d'une dissuasion nucléaire et de la capacité de mener des opérations de haute intensité. Pour demeurer dynamique, cette relation spéciale doit être nourrie de réalisations concrètes, d'opérations conjointes. » cet amendement a pour objet de rappeler que, dans la perspective d'un renforcement et d'une montée en puissance des coopérations européennes, le travail que l'on pourra réaliser avec le Royaume-Uni restera essentiel, notamment s'agissant de l'innovation et du matériel du futur. Quel Il revenait, bien sûr, à Mme Conway-Mouret de défendre cet amendement, qui tend à souligner l'importance de la coopération avec le Royaume-Uni. Je pense que nous partageons tous, malgré la situation un peu délicate liée au Brexit, la volonté de poursuivre, en matière de défense et de sécurité, une coopération étroite

Pour maintenir les capacités d'intervention aéronavale de la France sur les océans, cet amendement tend à prévoir la possibilité d'engager des études pour le renouvellement, non pas d'un, mais

prématurément ; il suffit de passer quarante-huit heures sur place pour voir les effets des climats très rudes et de l'usage intensif que nos armées font de ces matériels. Il est absolument nécessaire

Un soutien accru doit s'accompagner d'un contrôle renforcé. Sur ce genre de marché, le contrôle passe par la publicité, et seule la transparence garantit le respect des règles. les règles sont celles du traité sur le commerce des armes que la France a ratifié au mois d'avril 2014. Ce traité implique des obligations. Ainsi, un État doit refuser un transfert de matériel militaire s'il a connaissance que ces armes pourraient servir à commettre un crime de guerre. C'est pour assurer le respect de ce traité que nous souhaitons renforcer le contrôle sur les exportations. Il existe déjà une procédure, mais celle-ci

Un contrôle pourrait réparer cette faiblesse. Il permettrait une réévaluation des autorisations d'exportations. L'objet de cet amendement s'inscrit en outre dans la démarche de nos collègues députés, qui ont renforcé ce contrôle parlementaire.

a déclaré qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France, laissant entendre que le temps des arrangements caractéristiques de ce que l'on a appelé la Françafrique était révolu. Je souscris à ce propos s'il signifie réellement une nouvelle approche de la relation entre la France et les pays africains. Or, pour construire cette nouvelle approche, nous avons besoin de confiance et de transparence. Tel est bien l'objectif de cet amendement, qui vise à renforcer le contrôle parlementaire sur notre politique de coopération militaire. Il faut savoir en effet que plus de 70 % de cette coopération est destinée à l'Afrique. Présenter un rapport au Parlement, c'est garantir plus de transparence, ce qui est un gage de confiance vis-à-vis des citoyens des pays africains. C'est aussi un gage de confiance pour la France, souvent accusée du double procès de l'ingérence et de l'abandon. Il s'agit également de prolonger les efforts déjà réalisés. Ainsi, la réforme constitutionnelle de 2008 a permis de faire ratifier les accords de partenariat de défense par le Parlement. Cette procédure souffre d'un manque de précision : ces accords formels fixent un cadre général qui ne précise ni le nombre ni le rôle des coopérants militaires français mis à disposition. Cet amendement vise à y remédier.

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées examine tous les traités, notamment les traités de coopération militaire qui interviennent entre nos pays. Elle a même la possibilité de nommer un rapporteur, qui peut procéder à des auditions et aller au fond des choses, dispositif qu'elle met en oeuvre régulièrement. En revanche, tout ce qui concourt à faire une publicité excessive

nous attendons que Mme la ministre nous aide à faire vivre le Sénat, tel qu'il vient de montrer sa puissance, sa capacité et sa volonté de servir l'intérêt national. Mes chers